Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 2 et l'annexe A, qui contient le tableau patrimonial de la sécurité sociale pour le dernier exercice clos.

Mme Laurence Cohen. Cet amendement tend à réaffecter à l'assurance maladie les dépenses engagées durant la pandémie et indûment affectées à la dette sociale. Le Gouvernement a décidé de faire porter en partie le coût du covid sur l'assurance maladie.

dans le cadre de ses programmes d'émission classiques, qui assurent les meilleures garanties de refinancement (moindre coût) et avec un horizon de très long terme de remboursement. La logique de ce raisonnement aboutit d'ailleurs à s'interroger sur la légitimité de la reprise d'une partie de la dette liée au covid-19 par la Cades, décidée en août 2020.

de l'Institut de recherches économiques et sociales (Ires), corroborée par les chiffres de la direction générale du Trésor, estime à 8,4 % du PIB le montant total des aides publiques reçues par les entreprises, c'est-à-dire 205 milliards d'euros en 2021

De plus, selon un rapport du Giec de février 2022, de 3,3 à 3,6 milliards d'humains vivent dans un contexte de fortes vulnérabilités liées au changement climatique. D'ici à 2030, jusqu'à 132 millions de personnes pourraient basculer dans l'extrême pauvreté en raison du changement climatique. En effet, si les pauvres sont ceux qui contribuent le moins à la crise climatique, ils sont aussi les premiers- et les plus durement Afin de respecter nos engagements climatiques, les sociétés françaises doivent accélérer leur transformation dans le but d'être plus respectueuses et plus résilientes au regard des risques sociaux et environnementaux. Cet amendement vise donc à rétablir l'article 3 du PLFSS en y ajoutant un alinéa 6 permettant de conditionner les aides aux entreprises à des contreparties sociales et environnementales qui devront être définies par décret.

de rétablir l'article 3 qui rectifie les tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse ainsi que l'objectif d'amortissement de la dette sociale pour l'année 2022. Cet article a été supprimé par l'Assemblée nationale en raison du rejet de l'ensemble de la deuxième partie du texte par les députés. Je suis bien évidemment favorable à ce rétablissement, car c'est un élément essentiel de la crédibilité de ce PLFSS. À travers ce sous-amendement, je propose de rectifier le tableau d'équilibre pour 2022 afin de tenir compte du rehaussement de l'Ondam de 0,6 milliard d'euros

les heures supplémentaires et le temps de travail additionnel, et de financer les efforts engagés au titre de la période hivernale, en particulier pour la pédiatrie. L'Ondam serait ainsi rectifié de 9,7 milliards d'euros par rapport au montant voté dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.

puisque cet amendement rétablit l'article en se fondant sur une pétition de principe selon laquelle les recettes pourraient être majorées du produit d'aides aux entreprises si celles-ci ne respectent pas des contreparties sociales ou environnementales.

Par ailleurs, un transfert de déficit cumulé à hauteur de 136 milliards d'euros a été voté en 2020. Cette reprise vise à financer dans les meilleures conditions qui soient les déficits cumulés non repris constatés au 31 décembre 2019, ainsi que les déficits des exercices 2020 à 2023 résultant de la crise sanitaire. Des recettes ont été affectées à la Cades afin d'assurer le remboursement de ces transferts, prévu au plus tard pour 2033. Supprimer ces recettes aurait pour conséquence directe d'empêcher le remboursement de la dette, ce qui serait contraire à la loi organique du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie. Il est pourtant essentiel de rembourser la dette sociale afin d'assurer la pérennité et la soutenabilité de notre système de protection sociale. Il y va de notre crédibilité financière.

très largement les hôpitaux et les autres établissements de santé dont les comptes sont déjà en déficit ou à peine à l'équilibre. Selon les fédérations hospitalières, les effets de l'inflation seraient évalués à plus de 1,1 milliard

Cet amendement vise à rétablir l'article 4 dans sa version adoptée à l'Assemblée nationale et à augmenter les financements des établissements de santé et du médico-social, afin de leur fournir pleinement les moyens de juguler l'inflation, sans pénaliser les personnes malades, en situation de handicap, en difficulté et les personnes âgées qui en dépendent. L'amendement

Face à cette situation, le Gouvernement fait l'autruche et renvoie les patients vers le 15 pour réguler l'entrée aux urgences des malades. Notre amendement vise donc à renforcer les crédits des hôpitaux pour 2022 afin de mieux couvrir l'ensemble des dépenses supplémentaires liées à la lutte contre le covid-19, à l'inflation et au rattrapage des soins qui ont été mis en suspens durant la pandémie. L'hôpital est en souffrance, mais également la médecine de ville et les établissements et services pour pour personnes âgées ! Nous sommes donc favorables à une augmentation des crédits de l'ensemble des sous-objectifs de l'Ondam. Cependant, pour garantir la recevabilité de notre amendement, nous préconisons une réduction des autres sous-Ondam. L'amendement

Il s'agit de financer les engagements pris pendant l'été et plus récemment qui visent à soutenir les établissements de santé, en particulier pendant la période d'épidémie hivernale.

ces crédits supplémentaires permettront de soutenir financièrement les agents exerçant la nuit et de faire bénéficier les puéricultrices et les aides-puéricultrices de la prime d'exercice en soins critiques qu'elles ne touchaient pas jusqu'à présent. La rectification de l'Ondam 2022 est ainsi portée à 9,7 milliards d'euros par rapport au montant voté dans la LFSS pour 2022.

Pourtant, ce soir vous déposez un sous-amendement visant à modifier l'Ondam rectifié en ajoutant 600 millions d'euros de dépenses, rien de moins ! Monsieur le ministre, le Gouvernement savait pourtant, depuis le mois d'avril, que l'Ondam serait largement dépassé- le comité d'alerte l'avait prévu et la Commission des comptes l'a confirmé en juin

dans le champ de l'assurance maladie s'élevaient, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, à 236,8 milliards d'euros. Ce montant a été révisé par le Gouvernement à 245,9 milliards d'euros dans le projet de loi de financement pour 2023, tel que déposé le 26 septembre dernier. Les surcoûts sont essentiellement liés à la crise sanitaire, avec les vagues occasionnées par les variants delta et omicron, en début d'année, mais pas seulement. Le contexte inflationniste inflationniste est également responsable d'une partie du dépassement. Ce soir, le Gouvernement a déposé un sous-amendement visant à ajouter 600 millions d'euros à l'Ondam rectifié.

avant que nous passions au vote. Surtout, je constate que, pour partie, il s'agit de prendre en compte des dépenses au titre de mesures effectives du 1 juin au 15 septembre. Pourquoi celles-ci ne figuraient-elles pas au sein de l'Ondam rectifié déposé le 26 septembre devant l'Assemblée nationale ? Quand nous parlons de sincérité des débats budgétaires, monsieur le ministre, ce ne sont pas des voeux pieux : il est indispensable que les textes présentés soient assis sur des hypothèses crédibles et justifiées. Sous ces réserves, et dans l'attente des précisions du ministre, la commission a, à ce stade, émis un avis favorable sur l'amendement de rectification du Gouvernement.

l'Ondam 2022. Je suis en accord avec cette proposition. Cependant, l'amendement vise également à modifier la répartition entre les sous-objectifs de l'Ondam pour augmenter les crédits des établissements de santé et prendre en compte l'inflation, à hauteur de 1,1 milliard d'euros. Or la rectification de l'Ondam 2022 que nous avions proposée dans le texte initial visait précisément à tenir compte du contexte d'inflation. Ainsi, elle comprenait déjà 0,8 milliard d'euros à destination des établissements de santé et médico-sociaux pour assurer la compensation de l'impact sur la charge non salariale d'une inflation nettement supérieure à celle qui avait été prévue lors du vote de la LFSS pour 2022. Ce complément de financement s'appuie sur une étude détaillée, dont les résultats ont par ailleurs été partagés avec l'ensemble des fédérations hospitalières. je rappelle que cette rectification de l'Ondam comprenait aussi 1,5 milliard d'euros supplémentaires, destinés à permettre le financement de la hausse du point d'indice dans les établissements de santé et médico-sociaux publics ainsi que des mesures salariales pour les salariés des établissements privés. Cette mesure découle elle aussi du contexte d'inflation particulier à cette année. contexte est donc déjà pleinement pris en compte dans la rectification de l'Ondam que nous vous avions proposée dans le texte initial. Nous sommes par ailleurs favorables à l'amendement de Mme la rapporteure générale qui rétablit l'article portant sur la rectification de l'Ondam, sur lequel je vais revenir.

émergé des différents groupes de travail du CNR, qu'ils soient territoriaux ou nationaux. Si le diagnostic est connu et partagé par tout le monde, il serait hasardeux de partir trop vite sur des solutions qui ont l'apparence de la simplicité. C'est malheureusement ce qui a été fait dans les années 1970 avec le ; nous en payons encore les effets. Cela explique donc ma prudence quant aux mesures à venir sur la restructuration de notre système. La parole

J'insiste, le dépôt du texte a eu lieu le 26 septembre, tandis que les mesures couvraient la période du 1 juin au 15 septembre. Ce n'est pas crédible. Surtout, si ce financement n'était pas assuré, pourquoi l'annexe 5 revendique-t-elle 200 millions d'euros à ce titre ? Les 370 millions d'euros au titre des mesures de l'été comprennent-ils ces 200 millions d'euros inscrits à l'annexe ou s'y ajoutent-ils ? En clair, les mesures Braun ont-elles coûté 570 millions d'euros ou l'annexe 5 était-elle fausse ? Enfin, comment se traduisent dans l'Ondam 2022 rectifié- celui que nous votons ce soir -les 400 millions d'euros que le Gouvernement a annoncés dernièrement à destination de la pédiatrie et des soins critiques ? Vous l'avez un peu évoqué, mais j'aimerais obtenir des réponses plus précises. Pourquoi seulement 186 millions d'euros sont-ils présentés à ce titre ? Surtout, on nous parle, pour financer en partie ces mesures, d'un fléchage du reliquat de la sous-exécution tarifaire pour l'hôpital et du dégel du coefficient prudentiel : est-ce à croire que ce qui était promis par le Gouvernement comme rendu aux hôpitaux est désormais fléché ?

du coût de l'alimentation, qui explose également et les touche très directement. Par ailleurs, dans le cadre des dépenses d'investissement, un certain nombre de ces établissements ont été retenus au titre des investissements dits « du Ségur », mais le coût des

Monsieur le ministre, vous bénéficiez d'une clémence particulière du Sénat aujourd'hui : il n'y a pas si longtemps, de telles modifications du budget de la sécurité sociale juste avant la séance publique avaient entraîné la suspension de nos travaux.

intervenir. Comme toutes les fédérations hospitalières nous l'ont dit, la dépense d'énergie est insuffisamment prise en compte. Ce n'est pas réaliste. Nous ne pouvons pas délibérer dans des conditions satisfaisantes. Bien sûr, votre sous-amendement est le plus favorable, mais nous ne le voterons pas, parce que nous n'acceptons pas ces conditions d'examen.

est à Mme la rapporteure générale. La loi prévoit que, dans le cadre de l'expérimentation du versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne, les clients de prestataires perçoivent directement de l'Urssaf le montant des aides Or un dispositif spécifique de versement immédiat des aides aux clients de prestataires a été créé par la LFSS pour 2022 afin de permettre aux Urssaf de verser directement au prestataire le montant des aides C'est par le biais de ce dispositif qu'a été mise en oeuvre la généralisation, en 2022, du versement immédiat des aides fiscales aux clients de prestataires. L'expérimentation devant être prolongée, cet amendement de coordination précise que le dispositif généralisé dédié aux clients de prestataires est utilisé dans le cadre expérimental.

L'avance immédiate est un dispositif nécessaire pour soutenir la trésorerie des salariés, l'accès à la garde d'enfants et la création d'emplois déclarés dans le secteur des services à la personne. Elle a été généralisée avec l'ambition d'inclure tous les acteurs et toutes les activités des services à la personne. Or le Cesu préfinancé est totalement absent du dispositif, excluant de fait ses 800 000 bénéficiaires et 1 million d'intervenants. Ce titre spécial de paiement permet aux employeurs, publics comme privés, de participer au financement des services à la personne utilisés par leurs salariés. Avec un volume de 1 milliard d'euros émis chaque année, il s'agit d'un avantage social clé dont les objectifs rejoignent ceux de l'avance immédiate la réduction du reste à charge des particuliers et la simplification des démarches permettent de mieux concilier la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, en particulier les travailleurs en situation de handicap, les aidants et les familles, et de réduire le recours au travail non déclaré. Près de la moitié des salariés bénéficiant de Cesu préfinancés les utilisent pour de la garde d'enfants. La persistance de l'exclusion du Cesu préfinancé du dispositif d'avance immédiate installe une inégalité entre les salariés aidés par leur employeur et les autres particuliers employeurs, à l'inverse de l'intention du Gouvernement, qui a justement accéléré l'élargissement à la garde d'enfants. Des solutions opérationnelles peuvent être mises en place rapidement, d'ici à la fin de l'année, afin de pallier cette carence et de garantir l'accès de l'ensemble des acteurs au dispositif.

Monsieur le ministre, cette disposition dans huit semaines, c'est-à-dire dès le 1 janvier 2023, nous semble prématurée. Le bénéfice d'un Cesu préfinancé fait partie des prises en charge qui nécessitent des développements spécifiques. Nous échangeons d'ores et déjà avec les émetteurs de titres en ce sens. Nous n'avons naturellement aucune opposition de principe à leur inclusion dans le projet, dès lors qu'une solution technique permettra de mieux identifier, au sein des Cesu préfinancés, les dépenses réellement exposées par le salarié, ce qui est

associées à un paiement en ligne de fournir aux particuliers employeurs les renseignements nécessaires à l'établissement des déclarations Cesu. Il s'agit ainsi de lutter contre le travail au noir, même occasionnel, voire involontaire, provoqué par un défaut de communication des renseignements nécessaires, et, ainsi,

dans la mesure où sont évoqués les prestataires de services, tandis que l'exposé des motifs mentionne les salariés du particulier employeur. En tout état de cause, les dispositifs Cesu et Cesu+ permettent de déléguer à l'Urssaf le calcul et, surtout, le recouvrement des cotisations sociales et du prélèvement à la source

l'amendement n° 704. Cet amendement a pour objet d'augmenter significativement la taxation des retraites chapeaux les plus importantes. Aujourd'hui, le taux de la contribution due par les bénéficiaires de rentes supérieures à 24 000 euros par mois-

%. Les retraites chapeaux sont des rentes viagères versées par les entreprises à certains salariés, les sommes ciblées ici concernant plutôt des cadres dirigeants. Ce dispositif est actuellement exonéré de cotisations sociales et de la contribution sociale généralisée

de cette annonce, notre amendement vise à revenir sur la fiscalité des sommes, parfois indécentes, que reçoivent les personnes concernées. En France, en 2020, les 17 millions de Français à la retraite percevaient en moyenne 1 500 euros bruts de pension par mois,

défendu. Quel est l'avis de la commission ?

Outre ce coût non négligeable pour les finances sociales, cette disposition concerne essentiellement des dirigeants et des salariés très bien payés de grands groupes.

La distribution de parts gratuites se substitue parfois à une politique classique d'augmentation des salaires, c'est-à-dire de rémunérations socialisées et fiscalisées, en privant ainsi de façon durable la protection sociale de ressources.

dysfonctionnement de la gestion des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif. La marchandisation de la prise en charge de nos aînés a ouvert boulevard à la spéculation financière et à ses dérives en matière de conditions de travail des personnels, de non-respect du droit syndical dans les établissements, de détournement de fonds publics et, enfin, de maltraitance des résidents. C'est inacceptable. Nous sommes favorables à l'interdiction

à but lucratif : rationnement de la nourriture et des fournitures médicales, transfert de charges entre sections au détriment des financements publics pour doper la rentabilité financière, pression sur le personnel, opacité quant aux profits tirés de la spéculation immobilière, etc. Alors

À l'issue des travaux de la mission d'information du Sénat, il apparaît que les taux de profit insolents de ces grands groupes privés à but lucratif, supérieurs à la moyenne du CAC 40, sont rendus possibles par des mécanismes de prédation appuyés sur les dotations publiques et par l'industrialisation de l'accompagnement des personnes âgées. Ainsi, sans aucune prise de risque, compte tenu de l'évolution démographique du pays, des profits sont engrangés au détriment des usagers et des contribuables, par le recours à l'optimisation fiscale. Par cet amendement, nous proposons de taxer à 8,55

il me paraît nécessaire de travailler avec les partenaires sociaux et les collectivités territoriales à l'identification des recettes potentielles de la branche autonomie, avant de mettre en place diverses contributions par voie d'amendement.

Cet amendement a quant à lui pour objet de créer une redevance applicable aux Ehpad dont l'autorisation d'activité par les pouvoirs publics prévoit un pourcentage de places habilitées à l'aide sociale inférieure à 50

par l'opérateur, lui permettant de financer principalement le salaire des soignants, à travers la section soins. Les opérateurs publics et privés peuvent donc en bénéficier. Les Ehpad qui ne sont pas majoritairement agréés à l'aide sociale peuvent fixer librement leurs tarifs sur la section hébergement,

Par ailleurs, la vraie question qui est posée est celle de la place du privé à but lucratif dans le système médico-social et des méthodes de régulation dont on use. Cette question relativement vaste appelle

Lubin. Cet amendement vise à créer une taxe sur les superprofits des grandes entreprises réalisant plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont le produit financera la branche retraite de la sécurité sociale.

Merci,

Le sujet peut paraître technique, voire austère, mais ses enjeux sont lourds en termes d'organisation de la protection sociale, de ressources humaines et d'accès au droit pour les assurés. Le projet d'unification du recouvrement des cotisations sociales remonte à la fondation de la sécurité sociale elle-même. À partir de 1952, les Urssaf se sont progressivement substituées aux caisses primaires de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales pour assurer la collecte des cotisations du régime général, les autres régimes généraux gérant eux-mêmes le recouvrement de leurs cotisations. Cette situation induisait une grande complexité pour les cotisants et une relative inefficience de la collecte. Compte tenu de la performance des Urssaf et des prérogatives prérogatives spécifiques dont elles disposent, notamment leur capacité de diligenter des contrôles sur pièces et sur place, le projet de leur confier le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales a progressivement émergé. Mais au-delà de la volonté, il faut des moyens. Notre rapport d'information

les données individuelles, de mettre en oeuvre des conventions préalables entre l'Urssaf et les organismes gestionnaires des réseaux et enfin d'assurer la normalisation des modalités de calcul et de recouvrement des cotisations sociales de tout régime de la sécurité sociale.

Nous contestons cette disposition, car elle revient à réduire la pénalité de celui qui a fraudé. Nous souhaitons qu'en cas de fraude sociale aux cotisations- la fraude

En outre, le recours à la sous-traitance est de plus en plus souvent dévoyé par les employeurs et employeuses pour se soustraire à leurs responsabilités et obligations sociales, juridiques, voire fiscales, avec pour objectif de réduire les coûts de production pour accroître les profits. Souvent, l'objectif est de contourner les statuts sociaux des salariés : recours abusif au temps partiel, précarisation des salariés à travers des clauses de mobilité punitives, conditions d'emploi dégradées et déresponsabilisation des donneurs d'ordre quant aux conditions de travail. Cet amendement vise donc à supprimer l'alinéa 9,

revenir sur le plafonnement à 15 000 euros pour une personne physique et à 75 000 euros pour une personne morale de l'annulation des exonérations ou réductions de cotisations sociales dont bénéficierait le donneur d'ordre ayant manqué à son devoir de vigilance en matière de travail dissimulé pour la première fois sur une période de cinq années.

est en effet fixé pour l'ensemble des donneurs d'ordre fautifs, qu'ils soient récidivistes ou non, à 15 000 euros pour une personne physique et à 75 000 euros pour une personne morale. Aux termes de l'article 6, ce plafond ne s'appliquerait plus qu'aux donneurs d'ordre commettant leur premier manquement sur une période de cinq années. Les autres ne bénéficieraient plus de ce niveau de plafonnement, mais se verraient infliger une annulation proportionnelle aux sommes mises à leur charge au titre de la solidarité financière à l'égard du cocontractant ayant commis l'infraction de travail dissimulé. Dans le souci d'intensifier la lutte contre la fraude aux cotisations sociales, j'émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements

préconisait de reporter l'unification du recouvrement, le Gouvernement accélère la mise en oeuvre de son projet. Alors que l'ensemble des organisations syndicales et patronales s'opposent au transfert des cotisations des régimes complémentaires de retraite, le Gouvernement n'en tient pas compte. La tentation est grande pour Bercy de mettre la main sur le pactole de 87 milliards d'euros de cotisations retraite des cadres et de remettre en cause les droits des futurs retraités. Cette nouvelle étape de l'étatisation de la protection sociale

à l'amendement de Mme Gruny, il vise à ce qu'une entreprise soit informée de la faculté dont elle dispose de demander la communication d'une copie des documents que l'agent chargé d'un contrôle auprès d'une entreprise appartenant au même groupe et sur lesquels il fonde ce contrôle. Bien que les entreprises concernées soient sans doute de taille suffisamment importante pour connaître leurs droits,

Chaque personne contrôlée est destinataire, dans le mois qui précède le début des opérations de contrôle par l'Urssaf, de la charte du cotisant contrôlé, qui lui présente l'ensemble du déroulement de la procédure de contrôle et précise les droits dont elle peut se prévaloir à chacune des étapes qui composent

Merci,

Or les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général doivent être en mesure de bénéficier du temps nécessaire pour effectuer leurs contrôles. Nous proposons donc d'abroger la limitation de la durée des contrôles dans les entreprises. La fraude est souvent réduite à la fraude sociale et, au sein de celle-ci, à la fraude aux prestations, qui n'en représente pourtant qu'un dixième- il est toujours intéressant de le rappeler. Cet effet de loupe vise à renforcer le contrôle social. Ne bénéficiant pas d'une telle attention, la fraude aux cotisations et la fraude fiscale sont incomparablement plus importantes. Alors que l'on chiffre son montant entre 80 et 100 milliards d'euros, la fraude fiscale ne bénéficie pas encore des moyens de contrôle qui permettraient d'en recouvrer une grande partie.

qu'à 13,4 milliards d'euros, ce qui signifie que des milliards d'euros échappent à l'État. Selon la direction générale des finances publiques, « la lutte contre la fraude fiscale est un enjeu majeur de souveraineté et de redressement des comptes publics et une condition essentielle pour faire respecter le principe d'égalité devant l'impôt devant l'impôt ». Dans un contexte d'accroissement des inégalités sociales, le juste contrôle des entreprises est donc primordial. Cet amendement vise à garantir aux organismes effectuant les contrôles le temps nécessaire pour les mener efficacement. La parole pour présenter l'amendement n° 812. Le 26 octobre 2022, la commission des finances du Sénat a publié un rapport d'information relatif à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Cette mission d'information devait tirer un premier bilan de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude. Nous regrettons d'ailleurs que la commission des finances du Sénat ait occulté le changement de philosophie du contrôle fiscal engendré par la mise en place de la loi Essoc du 10 août 2018.

alors que le montant de la fraude patronale est estimé par la Cour des comptes à près de 25 milliards d'euros. Dès lors que les entreprises n'ont rien à se reprocher, il n'y a pas de raison de limiter la durée des contrôles. La limitation des contrôles à trois mois contribuera à accroître les difficultés pour les inspecteurs de la sécurité sociale,

cette limite aux entreprises de moins de 20 salariés, en plafonnant à trois mois la durée des contrôles. Dans le cadre de l'expérimentation menée entre 2018 et 2021, il semble que 38,5 % des contrôles diligentés ont duré moins de trois tandis que les autres ont été prorogés. De plus, il convient de noter que la limite de durée n'est pas applicable dans certaines situations problématiques, notamment en cas de travail dissimulé, d'obstacles à contrôle ou d'abus de droit.

à la demande de l'entreprise ou de l'Urssaf. Cette limitation est acceptable pour des entreprises de cette taille, dans la mesure où les contrôles n'y revêtent pas les mêmes enjeux que dans les grandes entreprises. Il ne paraît pas souhaitable de limiter la durée des contrôles dans les entreprises de plus grande taille, où les sommes en jeu sont beaucoup plus importantes et la complexité des contrôles supérieure. Il s'agit en effet de garantir aux agents des Urssaf, un temps nécessaire à l'accomplissement de leur mission, de leurs contrôles et de leurs vérifications, ce que ne permettrait sans doute pas la fixation d'un délai limite de six mois

? L'avis est favorable sur cet amendement qui vise à contraindre les employeurs qui dirigent ou qui ont dirigé une entreprise éphémère à procéder sans délai à la transmission d'une déclaration sociale nominative aux administrations et organismes collecteurs des cotisations et contributions sociales qui en font la demande. En effet, il s'agit d'éviter le non-versement des cotisations et contributions sociales dues par ces employeurs lorsqu'il existe des présomptions graves et concordantes qu'ils ont contrevenu, qu'ils contreviennent ou qu'ils contreviendront à leurs obligations à l'égard de ces administrations et organismes,

liées aux entreprises éphémères. Aucun des indices prévus ne constitue en réalité un critère fiable, à lui seul, pour présumer de la fraude, surtout si l'on n'en retient que trois sur cinq. La problématique du repérage des sociétés dites « éphémères » est bien prise en compte par le Gouvernement qui, précisément, a souhaité faciliter les contrôles par une identification précoce des sociétés potentiellement frauduleuses. Pour gagner en efficacité, l'article 41 du projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit que les greffiers des tribunaux de commerce pourront transmettre des informations aux agents des organismes de protection sociale ou aux agents de l'État qui sont compétents en matière de fraude sociale.

Sans doute conscient des risques que présente ce projet pour les droits à retraite complémentaire de vingt millions de salariés, le Gouvernement propose désormais de le reporter d'une année supplémentaire. De fait, les Urssaf ne sont pas en mesure d'assurer, comme le fait l'Agirc-Arrco, la fiabilisation des déclarations des employeurs, salarié par salarié, ce qui se révèle particulièrement problématique dans le cadre d'un régime par points comme l'Agirc-Arrco, où le premier euro cotisé ouvre autant de droits que le dernier. ailleurs, l'unification du recouvrement social ne se justifie plus, dès lors que le projet d'instauration d'un système universel de retraites géré par une caisse unique a été abandonné par le Gouvernement.

et consignations (CDC) au titre des cotisations dues à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec), au régime additionnel de la fonction publique (RAFP) et au Fonds pour l'emploi

l'avis du Gouvernement ?

Merci, monsieur le ministre, de faire allusion à un rapport fort intéressant

Mme Pascale Gruny. L'article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale dispose qu'à l'issue d'un contrôle de l'Urssaf, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi d'une mise en demeure ou d'un avertissement. La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant, reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, sauf exceptions énumérées dans le code. Pour répondre aux observations de l'organisme de recouvrement, le cotisant dispose de trente jours, éventuellement renouvelables une fois, s'il le demande. Or, il vient d'être jugé qu'« aucune disposition légale ne contraint l'Urssaf à mentionner dans la lettre d'observations la possibilité pour la personne contrôlée de solliciter un délai complémentaire pour répondre auxdites observations ». Il est donc souhaitable que le cotisant soit informé de cette possibilité de renouvellement des trente jours. Quel est l'avis de la commission ?

: La parole est à M. Jean-Jacques Michau. Cet amendement a pour objet de pérenniser le système spécifique d'exonération de cotisations et de contributions sociales patronales pour l'embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi du secteur agricole. Pour rappel, ce dispositif est intéressant, car il permet aux employeurs qui embauchent des travailleurs saisonniers de bénéficier d'une exonération totale des cotisations patronales, pour les rémunérations inférieures ou égales exonération dégressive au-delà de ce seuil pour devenir nulle à hauteur de 1,6 Smic. Il permet chaque année la conclusion de plus de 900 000 contrats avec un montant de cotisations réduit. Chaque année, à l'occasion du PLFSS,

concernés. Dans un contexte de dumping social des concurrents européens de notre pays, notamment l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne, dans les filières de la viticulture, de l'arboriculture, du maraîchage, de l'horticulture, des pépinières viticoles, des semences le dispositif permet chaque année la conclusion de 900 000 contrats. Ainsi, pour continuer à produire en France, avec des standards sociaux élevés,

activité depuis maintenant deux ans. Nous finançons aussi le chômage partiel, le fonds de solidarité, les reports et exonérations de cotisations sociales durant la crise de la covid-19 ...

les Etarf avait pour objectif de favoriser l'embauche de salariés en CDI, dans la mesure où l'activité diversifiée de ces entreprises, auprès d'exploitants agricoles, de particuliers, de collectivités de collectivités territoriales ou d'entreprises privées justifiait plutôt le recours à des salariés permanents. Toutes les entreprises de cette catégorie n'ont pas une activité diversifiée, puisqu'elle englobe également de simples entreprises de travaux forestiers

rectifié . L'embauche d'un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et des contributions sociales à la charge de l'employeur dont le champ

et du paysage dans le champ de cette exonération. Exclues de la loi de finances pour 2015, ces entreprises bénéficieraient ainsi d'un coup de pouce fiscal estimé à 30 millions d'euros, un montant peu élevé pour les finances de l'État, mais extrêmement important au regard de la situation de ce secteur. Comme beaucoup après avoir souffert des conséquences économiques de la crise sanitaire, il connaît de nouveau des difficultés liées aux pénuries et hausses des prix actuelles.

pour l'embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi du secteur agricole, en passant d'un seuil de dégressivité de 1,2 à 1,25 Smic, ce qui permettrait de mieux prendre en compte la réalité des rémunérations des salariés concernés. Dans un contexte de dumping social des concurrents européens de notre pays, notamment l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne, dans les filières de la viticulture, de l'arboriculture, du maraîchage, de l'horticulture, des pépinières viticoles, des semences et de la polyculture, le dispositif permet, chaque année, la conclusion de plus de 900 000 contrats

Fialaire. Actuellement, les agriculteurs ont le choix entre deux méthodes de calcul pour leurs cotisations sociales : l'assiette triennale de droit commun, qui permet de lisser les revenus sur les trois années antérieures, ou l'assiette optionnelle, qui permet de cotiser sur les revenus de l'année précédente. Le changement climatique est une réalité. Les agriculteurs sont les premiers à en subir les conséquences. Ils doivent faire face à l'augmentation de la fréquence et de l'intensité d'événements climatiques défavorables. Lorsqu'ils subissent de graves intempéries climatiques, les agriculteurs qui choisissent l'assiette optionnelle sont fortement pénalisés par un calcul qui ne correspond pas à la réalité de leurs revenus. de l'amendement proposent de prendre en compte les revenus réels de l'année, sur la base d'une assiette provisoire, ce qui permettra aux agriculteurs d'affronter les difficultés.

intercommunale (EPCI) sont amenés à gérer des services d'aide et d'accompagnement à domicile, participant ainsi aux politiques de maintien à domicile et d'action sociale. Or les EPCI ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale

EPCI peuvent gérer les services d'aide à domicile dans le cadre d'un

Le présent amendement propose la mise en place d'un dispositif d'exonération transitoire des cotisations sociales des employeurs de la fonction publique sur l'ensemble des couvertures de protection sociale complémentaire. Ce mécanisme transitoire sera mis en place pour la période allant du 1janvier prochain aux dates respectives d'entrée en vigueur des dispositifs pérennes de protection sociale complémentaire en santé, pour les trois versants de la fonction publique. La disposition s'arrêtera au plus tard le 1 janvier 2026. Alors que l'ensemble des employeurs de la fonction publique doivent désormais obligatoirement participer au financement de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires, l'amendement a pour objet de garantir un haut niveau de protection en santé de ces derniers. Il s'agit d'assurer l'équité de traitement et le respect du principe d'égalité entre les agents publics. l'amendement n° 203 rectifié . Le présent amendement propose la mise en place d'un dispositif d'exonération transitoire des cotisations sociales des employeurs de la fonction publique sur l'ensemble des couvertures des couvertures de protection sociale complémentaire. Ce mécanisme transitoire sera mis en place pour la période allant du 1janvier prochain aux dates respectives d'entrée en vigueur des dispositifs pérennes de protection sociale complémentaire en santé, pour les trois versants de la fonction publique. La disposition s'arrêtera au plus tard le 1 janvier 2026. Alors que l'ensemble des employeurs de la fonction publique doivent désormais obligatoirement participer au financement de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires, l'amendement a pour objet de garantir un haut niveau de protection en santé de ces derniers. Il

qui constitue objectivement la formule permettant la plus grande mutualisation des risques sur une base solidaire. Il paraît donc opportun de réserver les avantages fiscaux et sociaux liés à ces cotisations, à des assurances souscrites dans le cadre d'un CCO, formule qui a sans doute vocation à se généraliser à l'avenir.

qui engagent au moins 15 % de leurs charges en dépenses de recherche et de développement. En effet, une interrogation triennale du dispositif permettrait d'en contrôler la bonne efficacité alors que le volet social du dispositif JEI ferait l'objet de près de 50 millions d'euros de fraudes ou de déclarations erronées chaque année. Quel est l'avis de la commission ? qui, d'une part, réserve aux lois de financement de la sécurité sociale le droit d'instaurer des niches sociales de plus de trois ans- le dispositif, dont il est question ici, a été créé par une loi de finances -et qui, d'autre part, prévoit une évaluation de chaque niche sociale sur une base

à l'Établissement national des invalides de la marine, de la cotisation d'allocations familiales et de la contribution de l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi pour un coût évalué à 46 millions d'euros en 2020,

qui s'ajoute à l'avantage fiscal de la taxe dite au tonnage. Chaque fois, le chantage à la compétitivité et à la concurrence est avancé. En somme, le capitalisme s'exonère du modèle social pour préserver les règles de son modèle. Si CMA CGM bénéficiait de l'intégralité

l'amendement n° 707 rectifié. Cet amendement vise à prévenir les risques d'épuisement au travail en instaurant un malus pour les entreprises n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle. Le syndrome d'épuisement professionnel, plus communément appelé burn-out, est un phénomène croissant dans nos sociétés contemporaines. Les chiffres de cette épidémie discrète sont alarmants : l'Institut de veille sanitaire évaluait en 2015 à près de 500 000 le nombre de salariés en état de souffrance psychologique liée au travail, parmi lesquels 7 % environ étaient en épuisement professionnel- il est évidemment très difficile d'obtenir des chiffres solides. Cet amendement tend donc à prévenir les risques d'épuisement professionnel en incitant les entreprises à prendre les mesures nécessaires pour éviter les risques d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Concrètement, il s'agit de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.

préconisait la mise en place d'un tel malus lié aux accidents du travail. Cette proposition a en outre été reprise par M. Didier Migaud, alors Premier président de la Cour des comptes, lors de son audition par notre commission des affaires sociales en 2018.

Il a en effet pour objet la sous-traitance, mode d'organisation du travail de plus en plus fréquent et qu'il convient de dénoncer. S'il est demandé au sous-traitant de veiller à la sécurité de ses travailleurs, le donneur d'ordre est également, en principe, soumis à l'obligation légale de veiller à l'organisation de la prévention des risques liés à la coactivité. L'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale prévoit d'ailleurs que la valeur du risque qui aide à calculer les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles doit être partagée entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. Cependant, les donneurs d'ordres tendent toujours plus à externaliser vers leurs sous-traitants les risques physiques et psychosociaux associés à un travail d'exécution. Cette tendance inquiétante est confirmée par un rapport de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques

ainsi qu'à des horaires pénibles. Ce même rapport explique également que plus l'activité principale du donneur d'ordre est éloignée du site d'exécution de l'activité sous-traitée, plus ces risques sont importants. Pour toutes ces raisons, la répartition du risque doit être rééquilibrée. Nous proposons donc logiquement, pour pallier ces conséquences nocives pour les travailleurs, que les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles soient augmentées pour les entités ayant recours à la sous-traitance lorsqu'une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité fixé par décret. Il est temps de dénoncer les entreprises qui ont souvent recours à la sous-traitance ; je pense en particulier, parmi les scandales récents et plusieurs luttes

Le code du travail prévoit cependant que le responsable de l'entreprise utilisatrice doit assurer la coordination générale des mesures de prévention des risques professionnels qu'il prend et de celles que prennent les responsables de toutes les entreprises extérieures intervenant dans son établissement. En cas de risques spécifiques liés à la présence de salariés de différentes entreprises sur un même site, les entreprises concernées doivent établir un plan de prévention. En outre, la Carsat

par cet amendement d'élargir aux Ehpad et unités de soins de longue durée (USLD) du secteur public la réduction pérenne de cotisations sociales dont bénéficient les seuls Ehpad des secteurs privés, lucratifs et non lucratifs. À la différence des établissements sociaux et médico-sociaux associatifs et commerciaux, le secteur public ne bénéficie pas, depuis 2019, de l'abattement de charges pérenne de 8 % de la masse salariale. Cela représente une surcharge d'environ 400 millions d'euros Cette différence de traitement pénalise les établissements médico-sociaux publics, qui accueillent la grande majorité des résidents les plus modestes. Il est donc inéquitable de les surtaxer.

faibles ressources, car ils pratiquent des tarifs d'hébergement inférieurs, en moyenne, de 600 euros par mois à ceux du secteur commercial, mais aussi du secteur associatif. Par ailleurs, les tarifs d'hébergement n'ont pas suivi l'évolution des charges ; depuis bientôt dix ans, leur hausse est systématiquement inférieure à l'inflation. Les abattements de cotisations sociales doivent s'appliquer aux établissements publics ; à défaut, ceux-ci se trouvent dans une situation de désavantage concurrentiel qui menace leur pérennité à terme. je vous remercie

d'exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines. En effet, la réforme mise en oeuvre en 2019 ne permet pas, en l'état, de répondre à l'enjeu de création d'emplois hautement qualifiés outre-mer dans le domaine des nouvelles technologies et de la recherche et développement. L'appréciation de la réalité des « projets innovants dans le domaine des technologies de l'information et de la communication », ainsi que du périmètre des « salariés principalement occupés à la réalisation

puis dégressive jusqu'à 2,5 Smic. Au vu de ces paramètres, il est donc approprié de bien concentrer ce dispositif sur son objet, c'est-à-dire sur les emplois concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants. La commission émet un avis défavorable

de faire bénéficier les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics d'outre-mer du barème renforcé du régime d'exonération de charges sociales patronales spécifiques applicables aux entreprises ultramarines pour une durée de deux années s'étalant du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2025. filière est dans une situation critique ; elle doit donc bénéficier d'un allégement temporaire du coût du travail afin de maintenir l'outil productif et de sauvegarder les emplois jusqu'à la relance effective de l'activité.

ans. Il est donc proposé de faire bénéficier les entreprises du BTP de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion du barème de compétitivité renforcée du régime d'exonérations de charges sociales patronales applicables aux entreprises ultramarines pour le paiement de leurs cotisations dues sur les années 2024 et 2025.

Toutefois, si les performances commerciales de l'hôtellerie en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion sont souvent comparables à celles que l'on observe en métropole, les professionnels de la filière font face, depuis toujours, à des déficits de compétitivité du fait de la lourdeur de leurs charges d'exploitation, qui pénalisent la rentabilité et la capacité à se rénover. Ainsi, la masse salariale représente 42 % du chiffre d'affaires des hôtels aux Antilles françaises et 40 % à La Réunion, contre environ 30 % en métropole et 14 % dans les îles des Caraïbes voisines des Antilles françaises. La faible rentabilité des structures hôtelières dans les Antilles françaises a conduit à une diminution du parc hôtelier de 45 % en Martinique et de 38 % en Guadeloupe entre 2000 et 2022.

Quel est l'avis de la commission ?